La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat. Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein

Autre remarque, s'il est exact que les salariés des quatre entreprises destinées à fermer sont relativement bien informés de la situation, tel n'est pas le cas

bois faiblement traités, avec un objectif d'utilisation de 80 % de déchets bois et de 20 % de charbon, ce projet, me dit-on, participerait à l'économie circulaire, alors que, à l'heure actuelle, une partie

Mais pourquoi limiter cette mesure aux seules centrales à charbon de l'Hexagone et ne pas inclure celles d'outre-mer ?

Si le Gouvernement considère que les centrales à charbon sont une ineptie pour l'environnement et qu'il faut les fermer, il faut y inclure celles qui sont situées sur les territoires ultramarins

à compter du 1 janvier 2022, dont celle du Havre. Comme nombre de mes collègues, je m'étonne de l'adoption aujourd'hui d'une telle disposition, dont les effets ont déjà été annoncés, tant aux élus locaux qu'aux décideurs locaux économiques, le 12 avril dernier au Havre

Comme le prévoit l'article 3, fortement amélioré par le travail remarquable de notre rapporteur Daniel Gremillet et les amendements d'Élisabeth Lamure, que j'ai cosignés, il est essentiel que la fermeture soit accompagnée d'une politique forte à l'égard des salariés, en l'inscrivant directement dans la loi et en affirmant le rôle central de l'État, à l'origine de cette fermeture. À cet égard, je voterai l'amendement du Gouvernement tendant la prise en compte dans les procédures d'accompagnement des personnels portuaires, notamment des ouvriers dockers. En effet, la fermeture aura des effets sur toute l'économie portuaire, avec un impact fiscal, économique et social.

Je me félicite de la pugnacité des élus locaux, des acteurs économiques et portuaires et de l'État pour faire aboutir ce projet, qui, lui, sera créateur de 750 emplois. De même, je salue l'engagement du Premier ministre d'augmenter d'un gigawatt par an

cette bonne nouvelle ne doit pas réduire notre vigilance quant à l'accompagnement social et économique de la fermeture de la centrale à charbon du Havre, ancrée dans notre paysage depuis plus de cinquante ans. La parole est à Mme Céline Brulin,

si nous nous privions de ces capacités de production, pour importer de l'électricité produite dans des conditions parfois plus détestables encore ! Par ailleurs, nous toujours une réponse à la question soulevée par Fabien Gay. Nous avons besoin d'un bouquet énergétique, non pas parce que, pour des raisons idéologiques, nous défendrions les uns et les autres tel ou tel type de production, mais parce que l'électricité ne se stocke pas.

mais j'estime que la date de fermeture imposée aux centrales à charbon ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt des salariés de ces centrales, ni celui des collectivités locales. Voilà pourquoi je propose,

d'un délai suffisant entre l'adoption du texte et sa date d'entrée en vigueur. La date proposée ici permet d'assurer la transition industrielle et l'accompagnement social des sites. Elle est cohérente avec la directive sur le marché intérieur de l'électricité, également utilisée comme référence dans l'article 3. L'une des quatre centrales se situe en Moselle, au coeur d'une région où tant d'entreprises ont été fermées, dans un passé parfois pas si lointain, et au coeur d'un bassin qui,

nécessiteront du temps pour produire leurs effets, surtout si elles sont ambitieuses. Madame la ministre, je vous demande d'entendre l'appel des territoires ! Quel est l'avis de la commission ?

Monsieur le rapporteur, je ne voudrais pas être désagréable, mais vous dépassez votre temps de parole. Je ne l'ai pas beaucoup dépassé durant toutes mes interventions précédentes,

Je me réjouis donc de voir que, sur ces travées, on partage largement l'objectif d'arrêt de ces centrales à charbon.

montre que la fermeture des centrales à charbon ne pose pas de difficultés, même dans des scénarios pessimistes, dans l'hypothèse d'une

en termes d'approvisionnement énergétique, et ceci en toute transparence, puisque les différentes mesures ont fait l'objet d'une communication publique.

affectés par la fermeture de ces centrales à charbon. Nous nous inscrivons donc bien dans une vision d'ensemble, incluant l'enjeu en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prise en compte de la sécurité de notre approvisionnement énergétique, l'accompagnement

Une décision est prise par l'État. Dans sa souveraineté, l'État décide ; dans sa souveraineté, l'État assume toutes ses responsabilités, madame la ministre ! À un moment, il faut être parfaitement clair.

Je veux rappeler que la France, en 2016, n'a investi qu'un peu plus de 5 milliards d'euros dans le développement des énergies renouvelables et, au risque d'être désagréable, j'indiquerai que, sur 37 milliards d'euros de recettes de la taxe carbone, seuls 7 milliards d'euros ont été fléchés sur la transition énergétique. Comme d'autres, j'avais exprimé le mécontentement de notre assemblée

a été avancée, c'est-à-dire 5 % du total de l'effort de recherche, soit à peine 0,04 % du PIB. Par conséquent, quand on décide, on met en oeuvre les moyens et, à côté de l'État,

l'environnement l'emporte sur tout. Et c'est une idée assez facile à faire passer là où les choses vont bien,

! Quand on est confronté soi-même à cette situation-là, croyez-moi, on ne la vit pas de la même manière, qui plus est

du tout celles dans lesquelles on s'apprête à fermer les centrales à charbon : elle a fermé du jour au lendemain, du jour au lendemain pour les salariés, du jour au lendemain pour les collectivités territoriales et du jour au lendemain pour leurs finances.

en préconisant, compte tenu de l'atteinte portée par la mesure aux exploitants des centrales, que le dispositif doive être subordonné à l'existence d'un délai suffisant entre l'adoption du texte et sa date d'entrée en vigueur.

centrales. Et, madame la ministre, cela donne une autre dimension à la responsabilité de l'État, à votre responsabilité.

Le Gouvernement s'est déjà engagé à ce que le plafond d'émission qui sera fixé permette à la centrale de Cordemais de continuer à fonctionner pendant les quelques heures par an qui seraient nécessaires,

dans certaines configurations, notamment en cas de nouveau retard- comme c'est aujourd'hui acté -dans la mise en service de l'EPR de Flamanville. En revanche, la précision apportée n'apparaît pas utile au regard des engagements pris. Elle ne viserait par ailleurs que l'une des conditions citées par RTE, et non pas, par exemple, la mise en service de la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau, qui est pourtant visée dans l'objet de l'amendement. Enfin, et c'est là, madame la ministre, que nous avons encore besoin de précisions, concernant le projet Ecocombust,

ces analyses ont mis en lumière le rôle particulier de la centrale de Cordemais dans l'approvisionnement électrique de l'ouest. Le Gouvernement ne souhaite pas introduire dans la loi

rendu public en avril dernier, RTE déclarait : « En particulier, l'analyse des problématiques de tenue en tension montre qu'il est nécessaire que la fermeture des deux groupes de charbon de Cordemais intervienne seulement une fois que l'EPR sera mis en service.

Avec cet article, le Gouvernement nous demande une habilitation à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures permettant la mise en place par l'État d'un accompagnement spécifique pour les salariés qui perdraient leur emploi du fait de la fermeture des centrales thermiques à charbon. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 9 indique que ces mesures « favorisent le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut ». Cet amendement tend à remplacer « favorisent » par « prévoient ».

la crédibilité de la transition énergétique dans les milieux populaires, qui sont frappés de plein fouet par la désindustrialisation.

Vous le savez, nous en attendons beaucoup, et je serais fort déçu que vous n'alliez au bout

Cet amendement vise à donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés par les mesures que nous venons d'évoquer. L'article 3 devrait dès à présent préciser certaines des dispositions qui seront développées dans l'ordonnance et prévoir un financement public du dispositif d'accompagnement des salariés. La

de la prise en compte du statut, quand ce sera possible, ou de la mise en place par l'État de cet accompagnement spécifique. Ce dernier point est d'ailleurs plus précis que la notion de « financement public

la publication de l'ordonnance relative à la mise en place d'un accompagnement spécifique destiné aux salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, le Gouvernement devra présenter au Sénat et à l'Assemblée nationale la mise en oeuvre des dispositions prévues dans cette ordonnance. Nous estimons pour notre part nécessaire que le Gouvernement revienne régulièrement devant le Parlement, afin de permettre à ce dernier de disposer d'un suivi régulier de la mise en oeuvre de ces dispositions.

cet article comporte des dispositions sociales relatives à la mise en place d'un accompagnement spécifique des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon. Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que la commission des affaires sociales

Toutefois, les biocarburants de première génération, ou agrocarburants, qui sont produits à partir de cultures traditionnellement destinées à l'alimentation, comme l'huile de palme, le soja ou le colza, posent des problèmes qu'il convient de prendre en compte. En premier lieu, ils entraînent une déforestation considérable, notamment au sein des dernières forêts tropicales, de l'agrandissement des surfaces cultivées. On sait pourtant l'importance de conserver nos écosystèmes, d'autant que les forêts constituent des puits de carbones essentiels et que les motifs de déforestation sont déjà bien trop nombreux. L'accaparement des terres conduit également à une mise en concurrence avec les usages alimentaires.

Nous proposons donc de favoriser une mise en conformité de notre législation avec ces engagements, ainsi qu'avec nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, en sortant les agrocarburants de première génération de la catégorie des biocarburants à compter du 1 janvier 2020. Quel Quel est l'avis de la commission ?

à partir de coproductions, ils favorisent l'indépendance énergétique et protéique de l'Europe, ils assurent le développement d'emplois en milieu rural et ils diminuent le recours aux carburants fossiles. Naturellement, il faut éviter une concurrence entre utilisations énergétiques et alimentaires des produits issus de l'agriculture et s'assurer du gain environnemental que doit représenter l'utilisation de produits agricoles en lieu et place des produits pétroliers. Les biocarburants font l'objet d'une obligation d'incorporation cadrée par le code des douanes ; le taux d'incorporation est limité à 7 afin de concilier ces différents enjeux. Ces carburants doivent par ailleurs respecter un critère de durabilité : il doit être démontré qu'ils ne proviennent pas de terres riches en biodiversité et qu'ils assurent une réduction des gaz à effet de serre par rapport à un carburant classique. En conclusion, il n'y a pas lieu d'exclure systématiquement les biocarburants de première génération des dispositifs

mais simplement de vraies solutions et de vraies chances que nous devons donner à notre pays, en lui offrant une indépendance énergétique plus forte. Or, grâce aux biocarburants,

c'est vertueux ! Il n'y a pas de concurrence entre les produits alimentaires et non alimentaires : ce sont les mêmes productions. C'est une chance formidable, qui nous permet d'être moins vulnérables en matière d'approvisionnement énergétique et qui fournit une solution réelle pour notre économie et, qui plus est, pour notre agriculture. Nous

écologique. Les grands écrans numériques qui ont fleuri ces dernières années sont l'un des éléments qui incarnent ces contradictions et ces aberrations de nos sociétés. Notre amendement est assez simple : nous demandons l'interdiction de ces dispositifs publicitaires numériques.

». Nous proposons donc de débattre de l'interdiction de ces dispositifs publicitaires numériques.

énergivore, et ils consomment beaucoup d'énergie : un seul panneau correspond à l'équivalent de la consommation d'énergie, hors chauffage, de trois familles. Alors que la France s'est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d'énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d'urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent par conséquent plus être autorisés. D'après RTE, les gisements de baisse de la consommation portent sur les usages liés à l'éclairage, au froid et aux technologies de l'information et de la communication. De plus,

constitue ainsi une véritable pollution. L'éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont, par exemple dans une ville comme Paris, les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être

six heures du matin dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, la possibilité donnée aux maires de prendre des dispositions similaires dans les agglomérations de taille supérieure et la possibilité déjà

de creuser davantage ces sujets, afin de mettre à plat ce qui est déjà interdit et ce qui est laissé à la main des maires, de rappeler les conditions de mise en oeuvre des interdictions qui existent déjà et de reprendre ce sujet après une véritable évaluation et une concertation avec les collectivités concernées. Le Gouvernement demande donc le retrait de ces différents amendements.

Les éclairages nocturnes n'ont aucune utilité et prennent part de façon substantielle à la pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes. Un arrêté du 25 janvier 2013 prévoit déjà de telles mesures, soit appliqué dans les faits. Il est donc proposé d'intégrer cette disposition dans le code de l'environnement afin de lui donner une dimension plus coercitive. La parole

prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité d'un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L'article L. 121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

si la totalité des 3,8 millions de bénéficiaires initiaux du chèque énergie demandaient à être équipés, le coût global du dispositif pourrait être de l'ordre de 272 millions d'euros. Par ailleurs, en 2019, le Gouvernement a porté à 5,8 millions le nombre de bénéficiaires du chèque énergie,

prévue par la loi au seul accès aux données en temps réel. Cela permettrait aux consommateurs vulnérables équipés de smartphones d'avoir l'affichage en temps réel de leurs données de consommation. La modification proposée permettrait parallèlement de rendre possible la fourniture d'un afficheur dédié, complémentaire pour les consommateurs ne disposant pas d'un smartphone, dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. En effet, les certificats d'énergie ne peuvent être accordés pour des actions mises en oeuvre au titre d'obligations législatives ou réglementaires. Quel est l'avis de la commission ?

: ils ont été ajoutés lors des débats à l'Assemblée nationale, autant par les députés que par le Gouvernement, procédant au rafistolage d'une volonté politique et budgétaire défaillante. La majorité de l'Assemblée nationale a bien failli spolier un grand nombre de nos concitoyens- en l'occurrence, les propriétaires -de 5 % de la valeur de leur bien immobilier ! Heureusement, devant la levée de boucliers, le Gouvernement a reculé. Cette affaire de séquestre est symptomatique d'une politique où se mêlent idéologie et impuissance ! En effet, faute de moyens financiers pour accompagner bailleurs comme locataires dans la rénovation énergétique- c'est bien là tout le problème -, on a imaginé

Assommés de taxes et face à des rendements locatifs faibles, les propriétaires peinent de plus en plus à dégager le budget nécessaire à une rénovation. À agiter séquestres et plafonnements en tout genre, que fait-on, sinon dissuader les investisseurs qui craignent l'instabilité législative, alors qu'un placement immobilier se programme bien au-delà d'une dizaine d'années ? Par-delà ce désaccord, nous partageons, madame la ministre, l'objectif de lutter contre les passoires thermiques et les logements indécents. C'est un problème climatique et énergétique, mais, plus encore, un problème social,

pour les inciter à rénover leur logement. Enfin, il serait urgent de simplifier ce millefeuille de subventions et de déductions accordées à l'échelon local, régional ou national, tout comme il serait bienvenu d'y voir un peu plus clair dans les multiples labels énergétiques et de qualité.

à moyen et à long terme, pour assurer le financement des investissements publics en faveur de la transition énergétique, notamment celui de la rénovation thermique des bâtiments ». En effet, l'État doit mener une politique beaucoup plus volontariste en faveur de la transition énergétique. Il est donc essentiel de mobiliser les financements à la hauteur des ambitions et des engagements de la France. Force est de constater que le contexte actuel, marqué par une extrême faiblesse des taux d'intérêt, y est particulièrement propice. d'ailleurs pas échappé aux grandes entreprises, qui, depuis quelques années, ont massivement contracté des dettes à dix ou quinze ans sur les marchés financiers pour profiter des taux d'intérêt très bas et utiliser sur le moyen terme les fonds ainsi levés. Nombreux sont les économistes qui, aujourd'hui, pensent qu'il faut profiter de ce contexte de taux bas pour réinvestir massivement dans la transition énergétique. C'est le cas de Jean Pisani-Ferry et, plus récemment, d'Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du Fonds qui appelle même le Gouvernement à sortir de l'obsession de la dette publique et à utiliser le levier de la politique budgétaire pour relancer la production et l'emploi. Il est de la responsabilité du politique de se donner les moyens d'accélérer fortement la transition énergétique, notamment, compte tenu des enjeux, d'agir sur le secteur de la rénovation thermique des bâtiments. Il y a donc urgence à résorber la précarité énergétique dans un contexte d'augmentation du prix de l'énergie. D'après l'Observatoire national de la précarité énergétique, 5,6 millions de ménages français éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement- ménages dont les dépenses d'énergie dépassent 10 % et qui sont souvent contraints de sous-chauffer leur logement. Par ailleurs, plus de 30 % des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G de leur diagnostic de performance énergétique, ce qui représente une consommation très supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par an et par mètre carré ; pour 400 000 d'entre eux,

fasse l'impasse sur cette question. À l'évidence, les lois existantes ne sont pas à la hauteur des enjeux. On peut donc se féliciter de ce que l'Assemblée nationale ait eu la volonté d'introduire ce volet dans

tout à fait claires. Lui confier un rôle plus robuste serait de nature à clarifier les choses et à donner un meilleur accès à l'ensemble de ceux qui souhaitent entreprendre la rénovation de leur logement, qu'ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants.

Permettez-moi de vous livrer l'analyse en juin 2015 de M. Jean-Louis Bertrand, directeur scientifique de Meteo Protect : « Les entreprises qui doivent maintenir une température constante sont également touchées. C'est le cas dans l'agroalimentaire, dans les centres commerciaux, ou encore pour les sociétés qui ont des serveurs informatiques qui doivent être refroidis. Le problème est le coût de l'électricité qui monte en flèche. Leur consommation électrique augmente lors d'épisodes de forte demande énergétique, alors que l'offre, elle, ne suit pas. Les opérateurs sont donc obligés d'aller chercher l'électricité là où il en reste et paient donc très cher.

L'article 3 C se focalise sur une notion plus quantitative visant à définir de manière objective les bâtiments énergivores. La commission émet

est à Mme la ministre. La rénovation énergétique des bâtiments nécessite une expertise et des moyens dont ne disposent pas toutes les collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats de distribution d'électricité peuvent à cet égard avoir des compétences et une expertise utiles pour leurs membres. Leur donner la compétence de prendre en charge les travaux de rénovation énergétique des bâtiments permettrait d'accélérer la dynamique de rénovation des bâtiments des collectivités. Tel est le sens de cet amendement.

pour le compte de leurs membres, des travaux en vue de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Cette mesure étant de nature à faciliter la rénovation des bâtiments des collectivités territoriales, la commission y est favorable.

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, classée F ou G dans le diagnostic de performance énergétique. De De nombreux logements souffrent d'une piètre performance énergétique. Ainsi, quelque 8 millions de logements sont de véritables passoires thermiques. Dans l'attente d'un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d'entre eux,

une réponse urgente aux familles qui louent et qui doivent supporter des charges de chauffage extrêmement importantes. Il n'y a pas de raison qu'elles continuent de payer des loyers assez élevés, alors que les propriétaires ne font aucun effort

de performance énergétique, en fonction d'un maximum de consommation d'énergie finale, mais il ne prévoit pas suffisamment de mesures permettant de défendre les locataires de passoires thermiques,

il importe tout de même de prévoir des mécanismes afin de contraindre les propriétaires à entreprendre les travaux de rénovation nécessaires. À cet égard, cet amendement vise à limiter le loyer de

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement partage bien sûr l'objectif de déployer l'ensemble des moyens pertinents pour améliorer la performance énergétique des logements, en particulier pour mettre fin aux passoires thermiques. À cet effet, l'article 3 permet effectivement, dans les zones tendues soumises à un encadrement des loyers, en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, que les adaptations qui sont accordées dans que les adaptations qui sont accordées dans ces zones en cas de travaux ou de sous-évaluation ne soient possibles que lorsque le logement est suffisamment performant d'un point de vue énergétique. Les différents amendements qui sont présentés ici visent à soumettre l'ensemble des passoires énergétiques à un plafonnement ou bien à un mécanisme d'encadrement et présentent de ce fait un fort risque d'inconstitutionnalité, en ce qu'ils portent atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.

Angèle Préville, pour explication de vote.

Au-delà de ce seuil, un logement serait considéré comme indécent et ne pourrait pas être mis en location. La parole

et la lenteur des progrès dans la rénovation thermique de l'habitat. Seules 40 000 rénovations complètes ont eu lieu l'an dernier, et 250 000 partielles, alors que les objectifs chiffrés rappelés dans le plan Climat sur la rénovation de l'ensemble des passoires thermique, soit 7 à 8 millions de logements d'ici à 2025, et sur un rythme annuel de rénovation des logements de 500 000 par an, dont 100 000 logements sociaux, en ciblant le 1,5 million de passoires thermiques habitées par des personnes aux revenus modestes. Il nous faut donc clairement changer d'échelle et permettre un maximum de rénovations performantes complètes, qui soient véritablement efficaces. Pour cela, comme le suggèrent de nombreux acteurs, il faut commencer par définir plus rigoureusement les critères de décence des logements ouverts à location. Il faut en particulier que le critère de performance énergétique soit précisé, en fixant un seuil de consommation maximale. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kilowattheures par mètre carré et par an en énergie finale.

Il s'agit d'inciter les propriétaires de ces logements à effectuer des travaux d'amélioration énergétique. Nous proposons de fixer un seuil de 330 kilowattheures par an et par mètre carré, afin de toucher davantage de logements de logements et d'inclure les catégories F et G des diagnostics de performance énergétique. La France compte entre 7 et 8 millions de passoires thermiques. Le Gouvernement avait proposé un seuil de 600 à 700

est à M. Éric Gold. Le droit en vigueur intègre un critère de performance énergétique minimale dans la définition du logement décent. Malheureusement, il demeure mal appliqué et il suffirait de déterminer par décret ses caractéristiques de manière plus exigeante que la seule référence à la présence présence d'une installation permettant un chauffage normal. L'article 3 du projet de loi modifie la loi du 6 juillet 1989, en précisant que ce décret doit désormais fixer un seuil maximal de consommation d'énergie primaire et finale à respecter pour considérer la décence d'un logement, au plus tard le 1 janvier 2023, soit dans trois ans et demi. Nous le savons, un logement mal isolé, souvent combiné avec des dispositifs de chauffage peu performants, pénalise les ménages les plus modestes, tant sur la facture énergétique que sur le confort minimal que l'on peut attendre Il y a donc urgence à renouveler le parc locatif : les propriétaires bailleurs doivent contribuer pleinement à cet objectif en rénovant leurs biens les plus énergivores qui leur assurent un complément de revenus. L'effort que nous leur demandons consiste simplement à atteindre la classe E au regard du diagnostic de performance énergétique. Le présent amendement vise donc à définir directement dans la loi un seuil maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents, applicable lors du renouvellement des contrats de location, et non aux contrats en cours. Les propriétaires bailleurs pourront ainsi profiter de la vacance de leur bien pour effectuer des travaux. Nous proposons que les logements les plus énergivores, soit les classes F et G, ne remplissent plus les critères de décence au plus tard en 2023. Si nous attendons jusqu'à cette date pour déterminer les critères de performance énergétique, nous estimons que les seuils doivent au moins exclure les passoires énergétiques.

la définition du logement décent et le rendrait moins lisible par les Français. Il convient par ailleurs de prendre en compte la situation spécifique de certains bâtiments,

est à Mme la ministre. La lutte contre les logements énergivores est une priorité du Gouvernement. La définition des logements indécents pour cause de consommation excessive en énergie est une première étape, sur laquelle pourront reposer d'autres dispositifs incitatifs pour la rénovation. Il est nécessaire que cette définition puisse être comprise par tous les ménages. L'ajout d'un critère en consommation d'énergie primaire complexifie significativement cette définition définition et induit un manque de lisibilité pour les citoyens. En effet, elle ne correspond pas à la consommation d'énergie perçue par les ménages, qui, eux, voient l'énergie finale. La consommation d'énergie

des conséquences dramatiques, puisqu'elle ferait sortir du parc locatif privé et social des millions de logements. La commission a déjà rejeté des amendements similaires et elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ces trois amendements

Le scrutin est ouvert.

Dans le même esprit que pour le précédent amendement, nous proposons de considérer explicitement dans la loi que les logements classés G au niveau de leur performance énergétique ne remplissent pas les critères de décence à compter du 1 janvier 2022, soit les logements dont la consommation est environ deux fois supérieure à la moyenne nationale.

est à Mme la ministre. Le présent amendement a pour objet, tout en conservant l'esprit de l'article 3 , c'est-à-dire la prise en compte de la performance énergétique du logement au titre de l'indécence, d'adapter ce critère aux règles particulières qui régissent les copropriétés. En effet, si des travaux de rénovation énergétique peuvent être effectués dans les parties privatives, l'essentiel des travaux qui peuvent être réalisés relève des parties communes et nécessitent une décision de l'assemblée générale. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter le dispositif de l'indécence pour le cas où le bailleur, en dépit de toutes les diligences qu'il aura accomplies, ne sera pas parvenu à faire adopter par le syndicat des copropriétaires les travaux à réaliser. Dans ce cadre, le présent amendement prévoit que le juge saisi par le locataire afin d'ordonner les mesures nécessaires à la mise en conformité de son logement ne peut ordonner des travaux de rénovation énergétique lorsque les seules mesures utiles relèvent de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Il ne remet pas en cause les autres droits attachés à la caractérisation de l'indécence des logements et assure ainsi un équilibre entre les différents impératifs en jeu. Quel est l'avis de la commission ?

sans politique sociale. Alors que le secteur du bâtiment représente à lui seul 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France, l'un des premiers chantiers qu'il convient d'ouvrir est celui de la lutte contre la précarité énergétique, qui touche près de 14 % des ménages. Derrière ce chiffre, il y a deux réalités : la première est d'ordre social, puisque 12 millions de citoyens sont dans la difficulté, voire l'impossibilité de pouvoir chauffer leur logement à un prix abordable. La seconde est d'ordre environnemental, au regard des 7,2 millions de logements français qui sont considérés comme énergivores. Sur le plan tant social qu'environnemental, il est inadmissible que près d'un Français sur cinq fasse l'épreuve du froid,

Nous tenons à rappeler l'engagement du Président de la République en faveur de la rénovation thermique des bâtiments, en soulignant néanmoins que, pour atteindre cet objectif, il faut nettement accélérer le rythme, et non reporter systématiquement les échéances. Nous souhaitons donc prendre acte de l'urgence climatique et sociale, qui alourdit à la fois notre facture carbone et la facture d'énergie de millions de Françaises et de Français. Par cet amendement, nous proposons que le niveau de performance énergétique devienne une condition à la location au plus tard le 1 janvier 2022, et non pas en 2023. Un an d'économie sur les charges, c'est une différence considérable pour les 5,7 millions de foyers concernés. Un an de diminution de notre empreinte carbone, c'est un investissement durable pour les 7,5 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète.

On essaie de nous expliquer que, en votant, cet amendement, on mettrait hors du marché des centaines de milliers de logements. Eh oui ! Pas du tout ! Je vous rappelle que l'indécence n'est pas l'insalubrité.

du logement décent donnée par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : il s'agit d'un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »

Ronan Dantec, pour explication de vote.

est là, notre problème ! Il faut donc absolument que l'on réussisse à définir entre nous, dans l'hémicycle, puisque l'on n'a pas eu le temps avant et que l'État ne nous a pas proposé de stratégie, une base de solution

Lienemann, pour explication de vote. Je constate que, quand les propriétaires sont pauvres, on ne peut pas faire. Et quand ils sont riches, on ne peut pas faire

soyons audacieux ! Nous souhaitons renforcer la définition du logement décent, qui est une bonne notion, mais insuffisante à notre avis. En théorie, un logement indécent ne peut pas être mis en location, mais nous savons tous que ce n'est pas la réalité. Certes, le locataire pourrait demander sa mise en conformité par voie amiable ou en saisissant la justice- dans le 93, il en aura pour une dizaine d'années ... -, mais, en zone tendue, le rapport de forces est tellement déséquilibré en faveur des propriétaires que les locataires utilisent rarement cette possibilité. Les locataires connaissent la lenteur de la justice, qui manque de moyens, et se trouvent en réalité captifs. Voilà la réalité Pis, ils ne peuvent même pas suspendre le paiement des loyers avec consignation à la Caisse des dépôts en cas d'inaction du propriétaire, cette faute étant considérée comme plus lourde que la non-rénovation thermique. Or, nous l'avons dit et répété, il faut maintenant accélérer le mouvement de la rénovation énergétique pour la planète, mais aussi pour les millions de locataires qui vivent dans ces passoires énergétiques et qui doivent choisir entre se chauffer ou payer leur loyer. À la précarité énergétique s'ajoutent donc une précarité économique et une précarité sanitaire, tant physique que psychique. C'est pourquoi nous reprenons cet amendement, qui avait été adopté en commission du développement durable à l'Assemblée nationale, et qui est un réel marqueur d'engagement.

et d'assurer sa cohérence avec la révision des objectifs de la transition énergétique, à savoir un objectif contraignant de 32 % d'énergies renouvelables avec des sous-objectifs d'augmentation annuelle des énergies renouvelables et récupération dans le secteur du chauffage et du refroidissement, ainsi que dans le secteur des réseaux de chaleur et de froid.

dont les enjeux énergétiques et écologiques sont particulièrement importants, notamment en milieu urbain.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement soutient cette proposition, qui traduit l'une des mesures discutées dans le cadre du groupe de travail que nous avons mis en place pour développer les réseaux de chaleur et la part de la chaleur renouvelable qu'ils fournissent. Les schémas directeurs des réseaux de chaleur étant très importants pour leur développement, il est pertinent de généraliser leur élaboration pour tous les réseaux de chaleur. Enfin, la question des réseaux de froid est également un enjeu majeur pour l'avenir et l'adaptation au changement climatique. Le Gouvernement est favorable

Je rappelle l'engagement du Président de la République de doubler le fonds chaleur. J'espère que, dans le cadre de la discussion budgétaire, la nouvelle ministre de la transition énergétique que vous êtes saura défendre cette position. Je mets aux voix